des parcours en santé (Étapes) est incontestablement une avancée dans la lutte contre les ruptures des parcours de soins, l'éloignement des soins et la désertification médicale. Pour un meilleur déploiement du dispositif, il apparaît important d'inscrire clairement à l'article 24 le principe d'interopérabilité sémantique, et non pas seulement technique.

L'objectif de l'amendement est donc satisfait. Par ailleurs, la notion de téléchargement de données structurées est restrictive et ne tient pas compte de la nécessité de garantir, dans certains cas, les exports sous format simple comme « date » et « taux de glycémie

M. Alain Milon. Le présent article prévoit les modalités d'entrée dans le droit commun des dispositifs de télésurveillance afin de garantir un financement pérenne de ces solutions.

pour deux raisons. Pour les utilisateurs des solutions de télésuivi, au vu du cycle d'innovation rapide de la filière du numérique en santé, un dispositif de radiation et de déremboursement progressif est susceptible de créer une forte instabilité

de la commission ? Cet amendement pose quelques difficultés rédactionnelles. Même s'il était corrigé, il tendrait à rendre facultative et à la discrétion de l'État, et non plus obligatoire, la réduction de la prise en charge d'un dispositif de télésurveillance est remplacé dans la liste de remboursement par un dispositif plus performant. Cette dégressivité automatique du remboursement d'un dispositif devenu moins performant a pour but de favoriser le recours aux dispositifs les plus performants

24, s'approche pour beaucoup de celui des dispositifs médicaux, il serait logique que la détermination du montant de la prise en charge soit discutée avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) et non fixée par arrêté ministériel. Quel est l'avis de la commission

Le problème est que le forfait de l'activité de télésurveillance doit rémunérer non seulement l'exploitant, mais également les actes et prestations du professionnel médical organisant la télésurveillance. Or les professionnels de santé ne prennent pas part aux négociations avec le CEPS. Il est donc nécessaire de maintenir une fixation du montant forfaitaire

cet amendement vise à prévoir explicitement la possibilité de scinder la base forfaitaire de rémunération de l'activité de télésurveillance, définie par arrêté, en deux parties : l'une rémunérant le professionnel de santé, de santé, l'autre l'exploitant ou le distributeur du dispositif médical numérique. Cette précision est de nature à préserver l'équilibre des relations financières entre ces deux parties, en évitant de faire de la prise en charge du dispositif une variable d'ajustement.

Les nombreuses expérimentations engagées depuis 2014 à travers le programme Étapes ont démontré que la télésurveillance pouvait être considérée comme un levier d'action permettant d'améliorer l'organisation des soins et de diminuer les dépenses de prise en charge. La télésurveillance s'impose comme une solution pour réguler l'accès aux soins et un outil d'aide à la prise en charge permettant la détection précoce des besoins par une communication facilitée.

Si la prise en charge a déjà été enclenchée, elle sera alors suspendue. En outre, il est rappelé que le niveau de prise en charge pourra être modulé, voire suspendu en cas d'inutilisation répétée du dispositif.

spécifiquement de subordonner la prise en charge à son utilisation effective. C'est une périphrase, mais elle signifie exactement la même chose. Vous souhaitez conditionner la prise en charge à l'accord du patient de transmettre ses données

permet de répondre à certaines difficultés d'accès aux soins, les pratiques doivent néanmoins être encadrées afin d'éviter certaines dérives. Les établissements mentionnés dans cet amendement bénéficient de dispositifs médicaux numériques de qualité,

et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé. Nous reviendrons, à compter de cette date, au droit commun de l'accord conventionnel du 14 juin 2018 sur la télémédecine. Cette convention prévoit déjà la possibilité pour tout médecin de recourir à la téléconsultation, quels que soient sa spécialité, son secteur d'exercice et son lieu d'exercice, en ville ou en établissement de santé- cabinet de ville, centre de santé, maison de santé, etc.

On connaît trop bien les effets pervers et destructeurs de la T2A dans les hôpitaux publics pour ne pas s'inquiéter de ses conséquences sur les établissements psychiatriques. Ce type de financement favorise la recherche d'actes rentables. À cet égard, les indicateurs retenus nous inquiètent : le nombre d'actes, de journées, de demi-journées, la durée du séjour, la file active, la qualité du codage, l'âge des patients, etc. De nombreux professionnels en pédopsychiatrie et en psychiatrie nous ont alertés. Selon eux, ces indicateurs vont automatiquement orienter les pratiques vers les actes qui permettent de recevoir de très nombreux patients, au détriment des soins de longue durée : consultations ponctuelles, programmes de courte durée, bilans divers, prescription de médicaments. Ces professionnels s'inquiètent du devenir des personnes qui ont besoin de soins intensifs, relationnels, pluridisciplinaires, au long cours, ajustés au plus près de leurs besoins. Nous partageons leur analyse. En effet, les soignants en psychiatrie ne sont pas là pour enchaîner les consultations et faire du chiffre. C'est déjà, précisément, ce qu'ils dénoncent au sujet de protocoles qui déshumanisent la relation avec le patient. C'est C'est pourquoi nous voterons de nouveau contre ces réformes de financement, qui nous paraissent totalement inadaptées et inefficaces pour notre système de santé. Je suis saisi

de permettre aux établissements concernés de disposer du temps nécessaire à l'appropriation et à la prise en main des nouvelles modalités de financement. Ainsi, les établissements resteront financés en 2022 selon leurs modalités actuelles, le dispositif transitoire actuellement en vigueur

La mise en oeuvre pleine et entière de la réforme du ticket modérateur est prévue au 1 janvier 2022 et ses modalités d'application relèvent du domaine réglementaire. Le ministère des solidarités et de la santé s'était engagé à publier le décret avant l'été 2021, mais le projet de décret ne semble toujours pas avoir été transmis aux fédérations hospitalières pour concertation. Une telle réforme nécessite des adaptations techniques d'ampleur, mobilisant divers acteurs, dont les éditeurs de logiciels. Le délai restant avant le 1 janvier 2021 ne paraît pas suffisant pour préparer et déployer les évolutions techniques nécessaires à l'entrée en vigueur de cette réforme au sein des établissements de santé. C'est pourquoi cet amendement vise à maintenir, de manière transitoire, durant l'année 2022, les modalités actuelles de financement du ticket modérateur, le temps que les nouvelles règles applicables soient clairement édictées et appréhendées.

Deux réformes majeures du financement des établissements sont engagées, l'une dans le secteur de la psychiatrie, l'autre dans celui des soins de suite et de réadaptation. Ces réformes lourdes ont été votées dans de précédentes lois de financement de la sécurité sociale ; il convient désormais de les mettre en oeuvre.

La commission avait entendu ces craintes. Nous avions émis des réserves dans notre rapport, avant, finalement, de choisir de faire confiance au Gouvernement sur ce point. Force est de constater que cette confiance n'a pas été honorée, puisque la commission a découvert, hier soir, après la discussion générale, cet amendement technique, qui vise à reporter l'application de la réforme nécessaire à 2023.

entre les différents acteurs. Il semble en outre préférable de séquencer ces réformes du financement des activités hospitalières et de disposer d'un délai supplémentaire pour la réforme du financement des activités de SSR.

Depuis plusieurs années, nous alertons le Gouvernement sur l'urgence de revoir le financement de ces établissements, notamment par la revalorisation des coefficients géographiques. Dans tous les départements d'outre-mer, les hôpitaux font face à des surcoûts liés à l'insularité, aux dépenses de personnel, aux frais d'approche- transports et taxes -, aux évacuations sanitaires, mais également à la mise aux normes des bâtiments en matière sismique et cyclonique. Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la sécurité sociale aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l'Hexagone de 26 % pour la Guadeloupe et la Martinique et de 31 % pour La Réunion et la Guyane, ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux. Ainsi, chaque année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée aux établissements de santé. C'est la raison pour laquelle, en vue d'assurer un financement réaliste et adapté à la situation des outre-mer, cet amendement tend à préciser les critères sur lesquels reposent les coefficients géographiques.

l'application de coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux, à l'exception de quelques forfaits. Si la situation des outre-mer est particulièrement préoccupante, la rédaction actuelle ne se trouverait pas améliorée par les précisions que tend à introduire cet amendement, lesquelles peuvent déjà être prises en compte

On le sait, les établissements de santé privés à but non lucratif participent pleinement au service public hospitalier, alors même qu'ils ne bénéficient pas d'une égalité de traitement tarifaire avec les établissements publics de santé.

un an ou encore la première naissance française d'un bébé après une greffe d'utérus de sa mère. La situation actuelle provoque une double inégalité de traitement, qui pèse sur les Espic : inégalité avec les établissements publics de santé, d'abord, puisqu'ils sont soumis aux mêmes contraintes et obligations de service public hospitalier avec des tarifs différenciés ; inégalité, ensuite, au regard des autres catégories d'employeurs de droit privé, qui font l'objet de financements publics, car ces derniers conservent le bénéfice des allégements de charges. Les Espic supportent donc un coût du travail plus élevé pour exercer leur mission de service public hospitalier. Cet amendement a pour objet d'alerter le Gouvernement sur les inégalités de traitement qui pèsent sur les Espic, acteurs incontournables de notre système de santé. Je sais, monsieur le ministre, que vous étiez très préoccupé par cette question

pour les établissements hospitaliers MCO s'est accompagnée de la dégradation de leur équilibre financier ». Je regrette, mais ce n'est pas vrai ! La T2A a eu un effet inflationniste, qui a entraîné une amélioration

non urgents. En réalité, si les malades consultent aux urgences, c'est en raison des pénuries de médecins généralistes et de la disparition des gardes le soir et le week-end. Nous avions déposé un amendement visant à rétablir l'obligation de garde

sont fortement liées. Un meilleur usage des services d'urgences par la population suppose une optimisation de l'offre de soins en ville, répondant à des demandes de soins non programmés qui doivent être pris en charge par les médecins libéraux ou salariés

cet amendement, qui porte sur les conditions de la contractualisation entre les services d'urgences et les professionnels en ambulatoire. Quel est l'avis de la commission ? L'amélioration de

aider leurs collègues aux urgences, en assurant des gardes ou des demi-gardes dans les hôpitaux, comme le prévoit d'ailleurs le code de la santé publique. Comme vous, je regrette qu'un précédent ministre de la santé, Jean-François Mattéi, ait décidé en 2003 de supprimer l'obligation des gardes en ville,

Ces amendements tendent à préciser que la dotation complémentaire attribuée aux établissements de santé sur la base d'indicateurs de résultats en matière de qualité et de sécurité des soins vient récompenser la lutte contre les erreurs médicamenteuses. Or la prévention des erreurs médicamenteuses fait bien partie de la sécurité des soins. Il existe ainsi déjà des indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui concernent la prise en charge médicamenteuse, comme le respect des bonnes pratiques en matière d'antibiothérapie ou la qualité du volet médicamenteux de la lettre de liaison. Par ailleurs, la Haute Autorité de santé a dressé en décembre 2020 le bilan des erreurs relevées dans la base des événements indésirables graves associés aux soins et en a tiré plusieurs recommandations à destination des professionnels et des établissements de santé. L'objectif des amendements semble donc satisfait par le droit en vigueur.

monsieur le ministre,

à plusieurs reprises sur les pratiques d'isolement et de contention dans les établissements psychiatriques et dénoncé leur caractère attentatoire aux libertés et à la dignité, comme le souligne régulièrement la Contrôleure générale des lieux de privation

le terrain et avec le sommeil des patients. Le fait d'associer et d'informer davantage la famille va également dans le bon sens, même si je regrette que notre amendement visant à informer les patients eux-mêmes de leurs droits ait été déclaré irrecevable. Mes chers collègues, au-delà des problèmes rédactionnels, nous devons nous interroger : pourquoi pourquoi de telles pratiques existent-elles encore et sont même en augmentation dans les établissements ? La raison est simple : les établissements psychiatriques manquent cruellement de personnel. Ces pratiques ne sont que la partie émergée de l'iceberg et n'existent que parce que les soignants n'ont pas d'autre choix.

Même si votre rédaction est désormais plus solide juridiquement, elle est inapplicable dans les faits, les soignants n'ayant pas les moyens d'effectuer ces contrôles. Telle n'est pas la conception qu'ils ont de leur métier.

qui s'appliquent à certains patients faisant l'objet d'une prise en charge psychiatrique. Il tire en cela les conclusions d'une décision du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021. En 2020, la crise sanitaire et les difficultés rencontrées par le Parlement pour légiférer tout au long de l'année

que des modifications législatives importantes devraient être apportées pour garantir le respect des droits et la dignité des patients, mais leur introduction dans ce texte lui paraît trop précipitée pour être réellement à la hauteur de l'enjeu. la hauteur de l'enjeu. Je rappelle que le PLFSS ne fait pas l'objet d'un avis du Conseil d'État, lequel serait pourtant particulièrement utile s'agissant de dispositions qui ont déjà été censurées à deux reprises par le Conseil constitutionnel, en juin 2020 et juin 2021.

J'avais déposé un amendement visant à favoriser la création d'équipes mobiles de psychiatrie et de pédopsychiatrie à l'échelle départementale. De telles équipes mobiles sont très importantes, très importantes, car elles pourraient intervenir à la demande du médecin traitant au domicile de patients psychotiques qui refusent de rencontrer un psychiatre

commission ? Le présent amendement tend à prévoir que le coefficient minorant les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation en vue de concourir au respect de l'Ondam ne puisse être différencié par catégorie d'établissements que pour tenir compte des allégements de prélèvements obligatoires dont peuvent bénéficier les établissements de santé à but non lucratif. De même, les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation, qui peuvent être différenciés par catégorie d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical, ne pourraient l'être que pour prendre en compte ces mêmes allégements.

les soignants passent leur temps à chercher des lits disponibles, des lits d'amont comme d'aval ; enfin, bien souvent, les patients restent des heures sur des brancards. Aussi, je ne peux m'empêcher de penser que ces hôtels hospitaliers participent, d'une certaine façon, à l'externalisation de nos capacités hospitalières et ce, à moindre coût.

Le renforcement de l'accompagnement financier des établissements de santé en vue de la mise en oeuvre de ces prestations, prévu dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, allait, me semble-t-il, dans le bon sens, au regard des freins identifiés lors de l'expérimentation lancée en 2015.

à des bénévoles. De manière générale, le recours aux agents « faisant fonction » s'est accru et la qualité de l'accompagnement s'est dégradée. Toute l'année, nous vous avons interrogés sur les « oubliés du Ségur à tel point que vous ne supportez plus cette expression. Depuis le mois de mai, vous prétendez avoir comblé des lacunes en application de l'accord de méthode conclu par M. Laforcade. Pourtant, six mois plus tard, les symptômes persistent : distorsion d'attractivité au sein du même secteur médico-social, dont certains personnels perçoivent le complément de traitement indiciaire (CTI) et d'autres pas 22 % des départs volontaires sont dus à cette distorsion. L'article 29 prévoit d'inscrire dans la loi que les professionnels de l'accompagnement oeuvrant dans des structures bénéficiant d'une prise en charge au titre de la sécurité sociale des autres établissements financés par les conseils départementaux, sans prise en charge, nous n'avons aucune visibilité. L'accord Laforcade renvoyait la question à une conférence sociale des financeurs, qui devait se tenir avant la fin de l'année : où en sommes-nous ? Nous aurions souhaité défendre des amendements visant à étendre le bénéfice du CTI aux sages-femmes des maisons de naissance, par exemple, ou au personnel des centres de santé, mais les règles en matière de recevabilité nous privent de ce débat, ce que nous regrettons. La parole est

Sur le fond, les négociations menées sous l'égide de M. Michel Laforcade avec l'ensemble des acteurs du secteur ont permis de compléter le champ initial du Ségur de la santé, qui couvrait les secteurs de la santé et des Ehpad. Les acteurs de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée

Ce rapport devra également comporter des recommandations pour parvenir à une harmonisation indispensable des rémunérations et des conditions d'emploi et éviter la pénurie que nous connaissons depuis au moins deux ans. En effet, le manque d'attractivité de certains métiers désorganise notre système de santé. Il crée des distorsions entre les établissements et les services publics et privés, particulièrement dans les zones rurales.

qui exercent les mêmes métiers, après avoir suivi les mêmes formations, ne perçoivent pas les mêmes salaires ? Les personnels ne le comprennent pas, nous non plus d'ailleurs.

et de réinsertion sociale, dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou encore dans une structure de la protection de l'enfance. Ces secteurs sont sinistrés. Ils doivent faire face depuis plusieurs années à de grandes difficultés de recrutement et à un turn-over important. La crise sanitaire amplifie le phénomène et épuise les professionnels ; certains quittent leur métier. Les associations gestionnaires sont confrontées à des fuites de professionnels d'un secteur à un autre et à une pénurie de personnel. De telles difficultés en matière de ressources humaines influent sur la continuité et la qualité des accompagnements, sur les prises en charge et sur le soutien à des personnes particulièrement fragiles et vulnérables. Cela peut aller jusqu'à des fermetures de lits ou de services. Face à une telle situation, qui est extrêmement néfaste pour les personnes accompagnées, il est nécessaire de prévoir les financements, afin de rétablir l'équité de traitement entre les professionnels, où qu'ils exercent et quel que soit leur statut. La parole

et des accords Laforcade sur l'amélioration de l'attractivité des métiers de la santé, du secteur médico-social et social, ainsi que les conséquences, positives ou négatives, sur l'offre de soins- cela vient d'être évoqué -, notamment dans les déserts médicaux. En outre, il tend à assurer au Parlement que les mesures salariales du Ségur s'appliquent bien à l'ensemble des professionnels travaillant dans les secteurs de la santé,

Comme nous le savons tous dans cet hémicycle, les difficultés et les fortes tensions en matière de ressources humaines influent sur la continuité et la qualité des accompagnements

La mesure est saluée, l'élargissement de la prestation de compensation du handicap (PCH) aux aides à la parentalité étant attendu. Pourtant, les modalités suscitent des interrogations. Le décret du 31 décembre s'applique dès le lendemain.

de juin, les départements ne pouvaient toujours pas procéder au paiement ! Résultat, après plusieurs mois de mise en oeuvre théorique, il est difficile de trouver un foyer ayant perçu la PCH Surtout, il est délicat d'affirmer qu'une telle aide répond aux besoins exprimés. Son versement est conditionné au bénéfice de la PCH aide humaine.

Notre pays va voir le nombre de personnes âgées de plus de 70 ans et 80 ans doubler d'ici à 2030 ou 2040. Pour chacun d'entre nous, la bataille est celle du maintien à domicile le plus longtemps possible. Cela induit évidemment une prise en charge de plus en plus complète et qualitative pour garantir l'autonomie de nos aînés. Vous nous proposez des ajustements paramétriques marginaux a besoin d'une refonte systémique ! Quels financements nouveaux mettez-vous en face de l'avenant n° 43 ? Une prise en charge à hauteur de 100 millions d'euros ! Or l'Assemblée des départements de France évalue le coût de la revalorisation à 600

et à l'allocation personnalisée d'autonomie garantit le principe du libre choix du mode d'intervention de la tierce personne à domicile. Le bénéficiaire de la prestation peut choisir entre trois modes d'intervention pour être accompagné à son domicile : le prestataire, le mandataire et l'emploi direct. Le secteur de l'emploi à domicile en emploi direct ou une structure mandataire est fortement concerné par les enjeux liés à l'accompagnement des personnes âgées et en perte d'autonomie. Les modes d'intervention en emploi direct ou une structure mandataire permettent de couvrir les besoins d'accompagnement des personnes âgées au plus près des territoires, notamment dans les zones rurales difficilement couvertes par ailleurs.

Il nous paraît difficile de voter un texte comprenant un volet autonomie qui occulte la moitié des acteurs accompagnant les personnes âgées ou en situation de handicap. C'est d'autant plus étonnant que le secteur est le premier concerné par l'avance immédiate du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile à partir du 1 janvier 2022. À l'instar de la création d'un tarif socle à l'article 30 pour les services d'aide à domicile prestataires, nous estimons nécessaire de définir un tarif de référence à l'échelon national pour les modes d'intervention du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

L'objectif est de réduire les disparités entre départements. Il faut améliorer la solvabilisation de l'offre des services en rapprochant les tarifs de leur coût de revient.

Ils permettent de financer des heures d'aide humaine, des prestations techniques et complémentaires. La mise en place d'un tarif plancher va, comme à Paris et dans tous les départements dont le taux APA horaire est inférieur à 22 euros, entraîner mécaniquement une diminution du plan d'aide pour les personnes au plafond, soit près d'un tiers des bénéficiaires à Paris. Actuellement, une personne en GIR 4 peut bénéficier de trente-quatre heures d'aide humaine, contre trente heures avec le tarif à 22 euros. Il y a donc deux solutions. La première serait de calquer le plafonnement sur celui de la PCH, à savoir un plafonnement en nombre d'heures. Toutefois, cela ne permet pas d'y intégrer des dispositifs techniques, qui ne sont pas quantifiables de la sorte. Une réflexion avait été menée sur le fait de dissocier les aides techniques et l'aide humaine. Mais cela nécessiterait certainement une réforme structurelle de l'APA, qui n'est pas forcément compatible avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'autre solution serait de relever les plafonds des plans d'aide définis à l'échelon national. Après, la question de la hauteur d'une telle hausse demeure. Aujourd'hui, la médiane de l'APA en France est de 20,45 euros. La fixation d'un tarif plancher à 22 euros représenterait une augmentation de 8 %.

est ainsi libellé : La parole est à M. le rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que le tarif plancher des services autonomie à domicile sera fixé non pas annuellement, mais tous les trois ans, afin de limiter la complexité de gestion, notamment pour les départements.

Le présent amendement vise à préciser qu'un délai maximum d'un mois est laissé au président du conseil départemental pour motiver sa décision de rejet, conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'action sociale

L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et administration encadre les délais de réponse de l'administration dans les cas de rejet implicite. Il prévoit notamment : « [ ...], à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront

à M. Bernard Bonne. Il a été démontré que les obligations imposées aux services non habilités au titre de l'aide sociale remettaient totalement en cause leur liberté tarifaire et leur équilibre économique. En effet, les prix sont fixés librement lors de la signature du contrat de prestation de service et évoluent ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie, compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services, en application de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles. et de moyens (CPOM) ne peuvent pas imposer aux services une diminution de leurs prix ni l'impossibilité d'appliquer le pourcentage d'évolution des prix fixés par arrêté interministériel. Le présent amendement, sans remettre en cause le principe d'une maîtrise de la participation financière des bénéficiaires, vise à encadrer les obligations qui pourraient être imposées aux services. L'amendement

l'encadrement nous paraît absolument nécessaire pour limiter le reste à charge. Ainsi que je l'ai indiqué, le public accompagné par les services à domicile, qui est un public vulnérable et en perte d'autonomie, doit être protégé. Il doit pouvoir accéder à des prestations d'aide et d'accompagnement à son domicile, quelles que soient ses ressources et partout sur le territoire national.

Dans un souci de simplification, le B du II de l'article 30 organise la transformation automatique des autorisations détenues par les actuels services d'aide et d'accompagnement à domicile en autorisations de services autonomie à domicile à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Il prévoit un délai de deux ans, à compter de la publication du décret mentionné au nouvel article L. 313-12-0 du code de l'action sociale et des familles, pour se conformer au cahier des charges des services autonomie à domicile qui sera établi par ledit décret. Cependant, un traitement différent pour les services de soins infirmiers à domicile est envisagé. Ces derniers seraient, pour leur part, tenus de déposer une nouvelle demande d'autorisation. Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette distinction entre les services. Quel est l'avis de

dire ! Nous avons effectivement privilégié l'efficacité et la rapidité, en introduisant dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale un certain nombre de mesures qui permettent de créer concrètement

le troisième alinéa de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui plafonne la participation de la CNSA au financement des dépenses induites pour les départements par l'avenant n° 43 de la convention collective de la branche de l'aide à domicile. En effet, ce plafonnement est calculé en proportion de la part des heures d'allocation personnalisée d'autonomie, de prestation de compensation du handicap et d'aide-ménagère assurées dans le département, par rapport au total des heures financées à l'échelon national, tous services confondus. été évoqué notamment lors des premières interventions. Ce plafonnement touche ainsi les départements dans lesquels l'offre des services associatifs est supérieure à la moyenne nationale. De ce fait, les départements sont proportionnellement moins financés, contrairement à l'objectif de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Il convient donc de supprimer ce plafond pour garantir un financement des départements proportionnel à leurs dépenses, sans modification du budget prévu par l'article 47.

Par cet amendement, je vous propose de corriger les effets pervers des modalités de financement des soins réalisés dans le cadre de la perte d'autonomie à l'échelle des territoires. Le financement des soins infirmiers réalisés au titre de la prise en charge de la dépendance est effectué selon deux modalités : soit à l'acte, sous le régime de la convention nationale des infirmiers, aux tarifs négociés, soit par convention, sous seing privé, avec des structures de type Ssiad. Dans le premier cas uniquement, les actes sont directement facturés à l'assurance maladie. Dans le second cas, l'inclusion des actes infirmiers dans les dotations Ssiad entraîne une sélection des patients pris en charge dans ces structures, au détriment, souvent, des patients diabétiques ou de ceux qui ont besoin de soins pluriquotidiens. C'est aussi un frein à l'égalité en matière d'accès aux soins. C'est pourquoi je propose l'externalisation du financement des soins infirmiers réalisés par le secteur libéral, dans le cadre d'une prise en charge conjointe avec les Ssiad, et la possibilité de les facturer directement à l'assurance maladie. Cette mesure a d'ailleurs fait l'objet d'une dérogation du 6 mars au 10 juin dans le contexte de la pandémie. Aujourd'hui, hélas ! les Ssiad et les infirmières libérales agissent en concurrence, alors qu'ils devraient intervenir de façon complémentaire.

en cas de couverture insuffisante par les conseils départementaux et la CNSA, notamment en raison de la hausse des cotisations patronales en lien avec cet avenant.

Même avis ! après-midi, la hausse historique des salaires des personnels des SAAD associatifs que cet avenant n° 43, que nous avons beaucoup évoqué, a permise. Permettez-moi également de répondre aux inquiétudes qui ont été exprimées sur l'effet de la hausse des cotisations patronales en lien avec cet avenant. Nous l'avons indiqué à de nombreuses reprises, mais je le redis aux départements comme aux employeurs : les financements de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale couvrent les hausses des salaires chargés.

présenté à l'article 30 , à savoir l'expérimentation d'une carte professionnelle pour les aides à domicile. Il s'agit ni d'une mesure cosmétique ni d'une question annexe : il existe aujourd'hui dix-sept intitulés de poste ou de diplôme pour une même réalité. Cela induit, d'une part, un éclatement des revendications sociales et, d'autre part, l'absence d'un statut de référence pour ces salariés. Cet article permettra également de faciliter le travail quotidien des aides à domicile : elles auront un accès garanti aux équipements de protection dans les pharmacies-

remis par les députées Monique Iborra et Caroline Fiat, met en avant un autre facteur d'inégalités : celui de l'éligibilité à l'aide sociale. En effet, seulement 12 % des places dans les établissements privés à but lucratif sont éligibles à l'aide sociale, contre 98 % dans les Ehpad publics. De plus, la crise sanitaire a mis en exergue la situation alarmante des Ehpad en France : manque de moyens, de personnel, risques psychosociaux et j'en passe ... Ainsi, pour assurer le bien-être de nos aînés et respecter leur dignité bien trop souvent

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement vise à soumettre les actions qui seront proposées par les Ehpad « ouverts » à l'accord du conseil départemental et de l'ARS, afin d'éviter les chevauchements de compétences et de favoriser la coordination entre tous les acteurs en charge de l'aide, de l'accompagnement ou du soin des personnes âgées. Il est important de favoriser la complémentarité des actions et la synergie entre ces deux instances.

L'article 31 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles les Ehpad pourront assurer une mission de centre de ressources territorial. Il n'apparaît pas utile d'inscrire dans la loi qu'un accord conjoint de l'ARS et du département est nécessaire.

dans celui de l'article 31, dont les modalités d'application réglementaires pourraient d'ailleurs tenir compte. L'opportunité d'en faire un article spécifique n'apparaît donc pas clairement. Je demande, sur ce point, l'avis du Gouvernement. Quel est l'avis l'avis du Gouvernement.

en raison des surcoûts liés à la pratique de la médecine dans ces zones. Cette majoration est aujourd'hui fixée par circulaire budgétaire. Inscrire son principe dans la loi permettra de renforcer la solidité des plans de financement des établissements ultramarins. Tel est l'objet de cet amendement. Quel Cet amendement tend à prévoir que l'objectif de dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux tienne compte de coefficients géographiques permettant de majorer les recettes des établissements et services en outre-mer en fonction de certains surcoûts d'exploitation substantiels et durables.

Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » Or il existe aujourd'hui un phénomène qui nuit à la bonne marche de la solidarité nationale : le non-recours aux droits.

manquent d'informations et sont découragées par des démarches administratives souvent trop complexes. Afin d'éviter le renoncement aux prestations, le présent amendement vise à informer toutes les personnes à partir de 65 ans de l'existence de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation personnalisée d'autonomie, afin de renforcer l'accès aux droits et de diminuer le non-recours. contribuerait à accroître l'effectivité des droits sociaux, que les services publics doivent garantir à l'ensemble des citoyens. Il éviterait à certaines personnes de se retrouver dans des situations encore plus complexes et de sombrer dans la grande pauvreté. Quel est l'avis de la commission Cet amendement vise à rendre obligatoire l'information de toute personne de plus de 65 ans sur l'existence de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

fortement demandées par les acteurs de terrain. En effet, la double tutelle de l'ARS et du conseil départemental sur les Ehpad hospitaliers pose aujourd'hui des difficultés.

il apparaît indispensable de faire le point sur les effets de cette double tutelle et d'identifier des solutions opérationnelles afin de remédier à ces défauts.

L'enjeu de l'égalité de traitement face au besoin d'aide et d'accompagnement à l'autonomie implique la suppression de cette barrière d'âge. Le code de l'action sociale et des familles prévoit que la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quels que soient l'origine

à savoir le conseil et l'accompagnement, qu'elle peut exercer aux termes de cet article auprès des services départementaux, en plus des MDA et des MDPH. Il tend donc à supprimer la possibilité pour la CNSA de jouer un rôle d'audit et d'évaluation,

est l'avis de la commission ? Dans 52 % des cas, la PCH est attribuée pour compenser les charges liées à un besoin d'aide humaine, mais la nouvelle convention collective des particuliers employeurs fait craindre une augmentation du reste à charge pour les particuliers en situation de handicap employant un aidant.

de la généralisation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne. Il est également sensible à la nécessité de garantir une plus grande équité entre toutes les interventions à domicile, quel que soit le statut du professionnel. Ainsi, dans la continuité de la mise en place d'un tarif plancher pour les interventions à domicile en mode prestataire, chargée de l'autonomie, s'est engagée devant l'Assemblée nationale à lancer un groupe de travail pour remettre à plat la tarification des interventions financées par les particuliers employeurs.

De plus, le calendrier a été initialement fixé sans tenir compte ni de l'ampleur de la réforme et des travaux que doit mener la HAS ni du faible niveau des ressources affectées.

toujours en cours d'élaboration, et de préparer leur prochain cycle d'évaluation ; d'autre part, de permettre aux organismes habilités de s'approprier les outils et méthodes d'évaluation développés par la HAS et de répondre au cahier des charges qu'elle aura défini. Quel

amendement vise à retarder cette entrée en vigueur au plus tard au 1 janvier 2024. Même si le référentiel d'évaluation de la qualité est toujours en cours d'élaboration par la HAS et si des évaluations des établissements ont dû être suspendues pendant la crise sanitaire, il ne nous semble pas pertinent de repousser l'application des nouvelles dispositions.

ainsi proposé de prolonger jusqu'au 1 janvier 2025 les autorisations des établissements qui n'ont pas communiqué les résultats des évaluations entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022. En conséquence, la commission est défavorable

Cet amendement vise à exclure les primes versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux Paralympiques du calcul du plafond de ressources d'attribution des différentes prestations sociales versées aux personnes en situation de handicap. Quel est l'avis de la commission Cet amendement tend à exclure les primes d'État versées aux sportifs médaillés aux jeux Paralympiques pour le calcul du plafond de ressources retenues pour le versement de prestations, comme la PCH ou l'AAH, ou pour la prise en charge des frais d'accueil dans un établissement social ou médico-social pour les personnes en situation de handicap.

pour se prononcer spécifiquement sur l'intérêt et le bénéfice du produit en fonction de leur connaissance du secteur. Cependant, cette adaptation peut ne pas être systématiquement nécessaire. Il nous semble qu'il convient plutôt de prévoir

par l'assurance maladie des dispositifs médicaux, ainsi que la possibilité de prise en charge par l'assurance maladie de dispositifs remis en bon état d'usage. Cette réforme répondait aux préoccupations des entreprises de l'économie circulaire- je pense notamment au réseau Envie précurseur en la matière -et visait à permettre la prise en charge par la sécurité sociale des fauteuils roulants d'occasion pour personnes handicapées, après remise en état correct de fonctionnement.

le projet de décret sur la nomenclature de la liste des produits et prestations remboursées au titre IV, qui concerne les véhicules pour personnes handicapées, c'est-à-dire les fauteuils roulants, inquiète les usagers. Deux menaces D'une part, le non-remboursement de fauteuils non sélectionnés par le référencement les ferait sortir des catalogues, des réseaux de distribution, voire du marché français.

spécifications techniques, qualité des produits et prestations, volumes nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant, etc. De même, elle a permis que certains dispositifs médicaux spécifiques, comme les fauteuils roulants, puissent faire l'objet d'une remise en bon état d'usage en vue de leur réutilisation par une personne différente.

Il s'agit d'une garantie bienvenue et je peux témoigner que c'est une demande forte de l'ensemble des associations du monde du handicap. La commission est donc très favorable à cet amendement.

il peut concerner divers types de dispositifs médicaux. Il serait donc un peu étonnant que la précision que vous proposez soit apportée uniquement pour le handicap et non pour les autres dispositifs médicaux.

Comme l'a rappelé ma collègue Laurence Cohen lors de l'examen de cette proposition de loi, ce sont majoritairement des femmes qui cessent de travailler pour devenir proches aidants. Il s'agit donc d'une mesure d'égalité sociale. L'amendement

de jours de congé dont peuvent bénéficier les fonctionnaires est fixé à 310 jours, dans la limite d'une durée de trois ans. Nous souhaitons permettre aux parents, à titre exceptionnel, lorsque la situation de l'enfant le nécessite, de bénéficier d'un renouvellement de congé sans attendre la fin du terme de la première période de trois

il lui paraît difficilement justifiable d'étendre le bénéfice de cette prestation aux seuls aidants de personnes atteintes d'un cancer, et non à ceux de victimes d'autres pathologies, qui sont d'ailleurs citées dans l'exposé des motifs. Je pense aux maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, qui peuvent tout autant nécessiter la présence d'un aidant. Je tiens par ailleurs à souligner que de nombreux dispositifs sont ouverts aux personnes atteintes d'un cancer qui ont besoin d'une aide en raison des répercussions de la maladie sur leur vie quotidienne. Sous certaines conditions, ces personnes peuvent avoir droit à l'APA ou à la PCH. Leur aidant peut être rémunéré ou dédommagé dans ce cadre, ou bénéficier du congé de proche aidant et de l'allocation journalière du proche aidant, Pour les enfants, les parents peuvent prétendre au congé de présence parentale et à l'allocation journalière de présence parentale. En outre, les proches de personnes en soins palliatifs et/ou en fin de vie peuvent quant à quant à eux bénéficier du congé de solidarité familiale et de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Enfin, la stratégie décennale cancer de février 2021 consacre, vous vous en souvenez probablement, une part importante à l'accompagnement des proches aidants, qui va bien au-delà d'un congé de proche aidant. L'amendement n° 168, présenté

proposons ainsi de créer une conférence nationale des générations et de l'autonomie destinée, à présent que tous les travaux préparatoires ont été rendus, à documenter les perspectives démographiques, médicales et socio-économiques du vieillissement et de la dépendance, donc les besoins des personnes âgées et des personnes handicapées, afin de « catalyser » les décisions relatives au financement des priorités qu'appellent ces constats. Le point crucial, vous l'avez compris, est le chiffrage. C'est en partie fait pour les personnes âgées,

de cette proposition de conférence nationale des générations et de l'autonomie qu'organiserait tous les deux ans le Gouvernement, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l'autonomie. Nous sommes sensibles, comme vous, à la nécessité de poursuivre la refondation des politiques de l'autonomie dans la continuité de la création de la cinquième branche. L'organisation, à échéances régulières, d'une conférence nationale qui réunirait l'ensemble des acteurs des politiques de l'autonomie favoriserait la construction d'une ambition forte pour le soutien de nos aînés et le renforcement de cette solidarité intergénérationnelle, une ambition partagée, concertée avec l'ensemble des collectivités publiques. création d'une telle conférence, monsieur le rapporteur, doit néanmoins s'envisager, nous semble-t-il, dans le cadre d'une refonte plus large de la gouvernance nationale et territoriale de l'autonomie. Il est impératif, en effet, que les orientations en effet, que les orientations fixées puissent être déclinées dans les meilleures conditions sur les territoires- je suis sûr que vous êtes sensible à cet argument -, ce qui implique notamment une réflexion sur l'articulation des compétences des différentes autorités chargées de les mettre en oeuvre. Cette réforme d'ampleur de la gouvernance des politiques d'autonomie constituera le troisième acte

nos concitoyens. Je vous propose de rejeter cet amendement de suppression.

à Mme la rapporteure. Il s'agit d'un amendement de clarification de terminologie en matière d'interopérabilité. L'expression « données structurées » peut faire référence, dans le domaine de la santé, à des formats d'interopérabilité avec des représentations complexes. Or, potentiellement, des exports simples, de type « date et taux de glycémie », peuvent être utiles. L'export interopérable de données peut emprunter deux voies : soit suivant des standards normés référentiels, rendus opposables par arrêté, soit par des formats potentiellement simples et pragmatiques. Cet amendement vise à maintenir ces deux approches de l'export interopérable, en substituant à l'obligation du téléchargement de données structurées celle de l'accès direct aux données.

que l'interopérabilité doit également être sémantique, en intégrant la notion de nomenclature. Cette nomenclature interopérable est au coeur du développement des systèmes d'information en santé. Il apparaît donc pertinent de faire ressortir la nécessité que les données collectées soient interopérables non seulement par leur format, mais également par la nomenclature utilisée.

est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement ?

en compte la vertu thérapeutique du produit et son apport pour le patient, traitant ainsi de manière distincte les produits à vocation curative et les produits de télésurveillance. La rémunération à leur juste valeur des thérapies numériques s'effectuera à volume constant,

fonction de leur valeur thérapeutique. L'article 33 prévoit ainsi déjà que, pour être présumé innovant, et donc être et donc être éligible à la prise en charge anticipée, le dispositif médical doit apporter des bénéfices cliniques ou des progrès dans l'organisation des soins, d'après les premières données disponibles.

il s'agit de prévoir que, en cas de refus du patient de la transmission par le professionnel de santé des données nécessaires à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation effective du dispositif médical numérique, celui-ci ne pourra

secrétaire d'État. Cet amendement de cohérence juridique tend à prévoir la possibilité d'appliquer des encadrements relatifs aux conditions de prescription, d'utilisation et de distribution pour les prises en charge dérogatoires des dispositifs médicaux,

parole est à Mme la rapporteure. Il paraît surprenant de calculer le montant de la pénalité, en cas de non-respect des engagements de l'industriel en matière de continuité des soins, sur le chiffre d'affaires réalisé au cours des vingt-quatre mois qui ont précédé la constatation du manquement, alors que la durée de la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques est limitée à un an non renouvelable. En conséquence, l'amendement vise à préciser que le montant de la pénalité sera calculé sur le chiffre d'affaires réalisé au cours des dix-huit derniers mois qui ont précédé la constatation du manquement, afin de tenir compte du fait qu'au-delà des douze mois de la prise en charge anticipée l'entreprise s'engage à mettre à disposition le dispositif médical numérique pour une durée complémentaire de six mois.

pour les continuités de traitement lorsque le médicament n'est pas inscrit au remboursement. En revanche, s'il s'agit de continuité de traitement alors que le produit est inscrit au remboursement, ce sont bien les conditions de prescription de droit commun qui s'appliquent. Quel est l'avis de la commission

fassent l'objet d'un état des lieux, d'un bilan et, le cas échéant, de mesures correctives. Le cadre législatif et réglementaire en France prévoit plusieurs dispositifs d'accès accéléré au marché, c'est-à-dire permettant aux patients d'accéder rapidement à des technologies médicales innovantes de manière temporaire et dérogatoire avant leur prise en charge dans le droit commun. Il s'agit notamment du forfait innovation, de la prise en charge précoce ou dérogatoire, de l'article 51 de la loi de financement de la Ces dispositifs sont complexes, tant en raison des conditions d'éligibilité que des procédures à suivre pour les dossiers, des exigences en matière de collecte de données et d'évaluation, des mécanismes de financement ou encore des conditions de prise en charge dans le droit commun. commun. Ils sont multiples et souvent exclusifs les uns des autres. Il est nécessaire de redonner de la visibilité à l'ensemble des acteurs du champ de la santé et de s'assurer de l'efficacité de ces dispositifs. Une évaluation globale globale doit également permettre leur mise en cohérence globale, au bénéfice de l'intégration maîtrisée, pérenne et efficiente de l'innovation dans le système de santé. L'ensemble des parties prenantes pourrait ainsi disposer d'une vision claire des mécanismes en vigueur et d'une analyse de leur pertinence. Quel est l'avis de la commission

que le Gouvernement remette au Parlement un rapport avant la fin de 2024- histoire de se donner un petit peu de temps pour écrire le rapport -, qui sera publié, bien sûr, et qui sera censé évaluer l'impact de la refonte des modalités d'accès et de prise en charge des médicaments innovants et analyser l'impact de la réforme

n° 355 rectifié. Le contexte de rigueur budgétaire et de réduction des déficits publics nécessite un effort de la part de l'ensemble des parties prenantes du secteur. cet effet, le Gouvernement envisage de faire davantage contribuer les laboratoires qui bénéficient de développements réalisés par leurs concurrents dans des indications données, lorsque leur produit est utilisé en association. J'y insiste, c'est un cadre bien particulier, des produits de laboratoires différents en association. L'objet de cet amendement est de contribuer davantage à l'efficacité budgétaire de la sécurité sociale en informant le CEPS

amendements identiques visent en effet à dispenser des remises prévues à l'article 34 au titre des « AMM miroir » les spécialités faisant l'objet de remises conventionnelles. Leurs auteurs partent ainsi du principe, comme certains industriels l'ont fait valoir, d'une prise en compte des utilisations en association

que vous proposez d'exclure du champ de cet article 34 ne nous semble pas pouvoir exister. Les médicaments visés à cet article ne font jamais l'objet d'un accord conventionnel pour les indications considérées. Pour résumer, je pense que vos craintes, si tant est qu'elles soient de cette nature, ne sont pas fondées, et que votre amendement est satisfait

Le périmètre des spécialités visées est imprécis et le cas des associations avec des médicaments biosimilaires n'est pas explicité. Enfin, l'introduction de cette disposition dans la loi est contraire aux principes du dialogue conventionnel. Au regard de ces éléments, nous proposons de renvoyer au cadre conventionnel, dont c'est l'objet,

l'avis de la commission sur ces deux amendements

La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article. Nous voterons cet article qui, pour une fois, correspond à l'une de nos propositions. En effet, cela fait plusieurs années que je lance l'alerte sur les pénuries de médicaments.

ou encore de la pharmacie centrale des armées aurait dû être fait plus tôt, afin de leur permettre de produire certains médicaments essentiels, Que de temps perdu, notamment pendant la crise sanitaire ! Selon notre groupe, c'est bien à la puissance publique de reprendre la main pour que nous retrouvions notre souveraineté sanitaire.

soit on continue à laisser les entreprises pharmaceutiques dicter leur loi et faire primer leurs profits, soit on se saisit d'outils publics pour répondre aux besoins des patients : de nombreux pays ont choisi

Trop imprécise, cette notion ferait peser une insécurité juridique sur les acteurs français, qu'ils soient hospitaliers ou industriels. Aussi, il est proposé de préciser la notion d'« absence de spécialité adaptée », afin qu'elle soit bien reliée à la situation médicale des patients.

par rapport à la notion d'« indisponibilité » déjà inscrite dans la loi pour les préparations magistrales et hospitalières. Cependant, l'étude d'impact montre que cette précision vise à permettre de recourir à ces préparations en cas de refus de prise en charge ou d'échec des négociations sur le tarif. Cette démarche va clairement au-delà des dispositions de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments

Aussi, nous proposons de supprimer l'ajout de la référence à une absence de commercialisation effective, afin d'éviter de faire entrer la France dans une voie contraire aux normes européennes. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements concerne l'amendement n° 97 rectifié, la notion de « spécialité pharmaceutique adaptée » renvoie à la situation médicale du patient. Ainsi, telle ou telle spécialité peut ne pas être adaptée à la prise en charge d'un enfant en bas âge parce qu'il est impossible d'en adapter la posologie.

Actuellement, certaines entreprises concentrent entre leurs mains les capacités industrielles de production de thérapies géniques. Celles-ci sont pourtant issues de la recherche financée par les fonds publics. Cet amendement, proposé par les associations Aides et Action santé mondiale, vise donc à autoriser la production par des structures hospitalières de ces thérapies géniques ou cellulaires.

d'autoriser les établissements publics de santé à produire des médicaments en cas de rupture de stock ou pour faire face à une menace. Nous avons bien vu pendant la crise sanitaire l'intérêt d'une telle possibilité, en particulier pour les produits de réanimation qui ont été ainsi fabriqués.

la base de négociation avancée par l'entreprise était de 1,8 million de dollars pour une thérapie à dose unique ! Les prix réclamés par les laboratoires sont aujourd'hui déconnectés des coûts

La production de médicaments de thérapie génique ou cellulaire fait l'objet d'un encadrement spécifique, compte tenu de leurs contraintes de production, ce qui explique que cette production n'est pas ouverte à toutes les structures hospitalières. En effet, ces médicaments entrent dans la catégorie des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, qui sont autorisés par l'ANSM. Les établissements et organismes autorisés à les produire doivent être habilités par le directeur général de l'ANSM. ont ainsi été autorisés à produire des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, qui comprennent notamment des produits de thérapie cellulaire. Cet encadrement est aussi une garantie de qualité et de sécurité pour les patients. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements

pour répondre à des ruptures de stock ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave. Il est prévu d'assurer le financement de ces activités par le biais des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Migac), conformément à l'intention du Gouvernement, inscrite dans l'étude d'impact, d'opter pour cette voie de financement. Le Gouvernement a en effet confirmé dans l'étude d'impact que « la mesure aura un impact sur les dépenses de l'assurance maladie par le biais du financement par dotation pour mission d'intérêt général qui sera versé aux établissements de santé concernés ». Il s'agit bien ici de sécuriser ce mode de financement.

Merci